Monsieur le Premier ministre, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, c'est avec émotion que nous avons appris le décès, lundi, de notre ancien collègue Nicolas Alfonsi, qui fut sénateur de la Corse-du-Sud de 2001 à 2014. Maire de Piana pendant trente-neuf ans, premier vice-président de l'Assemblée de Corse, premier vice-président du conseil général de la Corse-du-Sud, Nicolas Alfonsi a été un acteur majeur de la vie démocratique et de la décentralisation en Corse. Il a été le défenseur passionné de son île, qu'il a servie également au travers de la présidence du Conseil des rivages de Corse et des responsabilités qu'il a assumées en tant que premier vice-président du Conservatoire du littoral. député de la Corse-du-Sud en 1973, en 1981 et en 1986 avant de devenir sénateur le 2 décembre 2001- date symbole -et membre du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, il est toujours resté fidèle à son idéal républicain et à sa tradition radicale. Pendant treize années à nos côtés, Nicolas Alfonsi a éclairé notre assemblée et la commission des lois, dont il était membre, par la finesse de son analyse, la rigueur et la subtilité de son raisonnement juridique, façonné par son métier d'avocat. Sa grande culture historique, marquée de sa passion pour l'épopée napoléonienne, son sens politique conjugué à son sens de l'humour

La grande intelligence, les réparties parfois mémorables, l'indéfectible esprit de justice, de solidarité et de fraternité de ce grand républicain, de ce grand Français, de ce grand Corse vont cruellement manquer. Au nom du Sénat, je souhaite exprimer notre sympathie et notre profonde compassion à sa famille, à ses proches, ainsi qu'au président et aux membres du groupe RDSE, auquel il a appartenu. J'ai une pensée particulière pour son épouse. Je vous propose d'observer un instant de recueillement.

en votre nom à tous, à assurer de notre soutien et de notre profonde reconnaissance tous nos compatriotes- en particulier les personnels soignants, en ville et à la campagne, personnels hospitaliers des secteurs public et privé, soignants, administratifs ou techniques, ainsi que toutes les équipes de secours -qui sont engagés depuis plusieurs semaines maintenant dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le Sénat salue leur détermination, leur disponibilité et leur dévouement face à une crise sanitaire exceptionnelle qu'ils affrontent en première ligne, dans des conditions particulièrement difficiles. Ils méritent toute notre gratitude. Leur attitude exemplaire rend d'autant plus indispensable, en ces moments critiques, l'effort de responsabilité et de discipline exigé de chacun. Je souhaite aussi rendre hommage à tous ceux qui, à leur poste de travail, assurent la continuité des services de la Nation. Qu'ils soient agents publics ou salariés du secteur privé ou associatif,

pour nos deux collègues que j'ai eus au téléphone ce matin et dont les nouvelles sont rassurantes, ainsi que pour le président Requier,

Mes chers collègues, les conclusions adoptées par la conférence des présidents réunie ce jour sont consultables sur le site internet a fixé l'ordre du jour des séances de cette fin de semaine et, au regard des mesures de restriction de circulation et de réunion en vigueur, elle a décidé de retirer de l'ordre du jour les débats de contrôle et les textes législatifs qui avaient été précédemment inscrits pour les trois prochaines semaines. Vous serez bien entendu tenus informés des conditions dans lesquelles nous reprendrons nos travaux et assurerons notre mission de contrôle de l'action du Gouvernement, qui est aussi une mission essentielle. En l'absence d'observations,

ministre, madame, messieurs les ministres, mes chers collègues, à cet instant, nous entendons rendre hommage au travail remarquable du personnel soignant qui est en première ligne pour sauver des vies, parfois dans des conditions dramatiques, comme actuellement dans le Grand Est. Nous avons aussi une pensée émue pour les malades et leurs proches. Je tiens également à remercier nos concitoyens qui respectent les consignes sanitaires : ces mesures extraordinaires sont contraignantes, mais absolument nécessaires. Nous saluons enfin l'engagement des pouvoirs publics, des services de l'État, mais aussi des élus locaux et des agents mobilisés au quotidien. Au Sénat, nous avons fait le choix de traiter au travers de nos questions les différents aspects de la crise, afin d'obtenir les réponses les plus complètes du Gouvernement. complètes du Gouvernement. Notre continent est à présent le premier foyer de la pandémie. Pour limiter la propagation du virus et éviter la saturation de nos hôpitaux, l'Union européenne a renforcé le contrôle de ses frontières, et certains pays membres ont fait de même. Seule une solidarité intra-européenne permettra de faire face à cette crise qui ne connaît pas de frontières. Aucun des pays membres de l'Union européenne ne peut cependant vivre de manière autarcique le marché unique doit donc continuer de fonctionner, mais avec précaution et contrôle. Les réponses des États membres doivent être coordonnées et cohérentes. La coopération européenne doit jouer en matière

de matériel de protection et par la mise à disposition de crédits significatifs pour financer la recherche sur le Covid-19 et trouver un vaccin. La troisième série d'initiatives vise à

Cette crise va porter un coup d'arrêt puissant, massif et brutal à notre économie une transformation puissante, massive et brutale de nos habitudes collectives de vie. Elle fait courir

des sceaux, comme le Gouvernement et l'ensemble de la population, nous avons pris la mesure du défi que représente l'épidémie de coronavirus pour notre pays, mais aussi pour l'institution judiciaire,

vont être matériellement rendues quasiment impossibles en l'état des moyens de notre justice, outre le danger de propagation que présenteraient ces mouvements, comme l'a déjà signalé l'Association des magistrats. Nos juridictions et nos établissements pénitentiaires ne disposent ni de matériels de protection pour les personnels et les auxiliaires ni d'équipements de visioconférence en nombre suffisant. Les parloirs sont suspendus.

Madame la sénatrice Goulet, je sais que vous êtes très attentive à la situation des établissements pénitentiaires, en particulier ceux de Condé-sur-Sarthe et d'Argentan. Sachez que, dans le cadre du projet de loi d'urgence, nous allons prendre des mesures

Les mesures générales de confinement récemment prises empêchent les familles d'accéder aux parloirs qui, de fait, ont été suspendus, mais les avocats

que nous pourrons compter sur les avocats pour assurer le respect des droits de la défense dans cette période exceptionnelle. Soyez assurée, madame la sénatrice, que tous les personnels judiciaires et pénitentiaires sont actuellement pleinement pleinement mobilisés pour assurer la continuité du service public de la justice et la sécurité de nos concitoyens, cela dans le respect des droits fondamentaux de chacun.

Dans l'immédiat et dans l'urgence, la priorité, pour le Gouvernement, est de faire en sorte que nous puissions passer la crise sanitaire, passer la crise sanitaire, en permettant aux entreprises de survivre à ce trou d'air et de conserver leurs salariés, c'est-à-dire leurs compétences, de façon à pouvoir ensuite

il faudra aider l'économie française à rebondir, aider l'ensemble du tissu productif à reprendre du muscle et à repartir de l'avant.

une guerre mondiale contre un ennemi invisible, et pourtant si présent, comme l'a justement dit notre président. Pour autant, la France n'est pas restée derrière sa ligne Maginot. Nous sommes passés à l'offensive avec, dès samedi dernier, la mise en place de mesures inédites. Devant la gravité du moment, nous avons entendu l'ordre de mobilisation générale du Président de la République. L'heure de l'affrontement est arrivée. Au front, nos médecins, nos infirmiers, nos pharmaciens et l'ensemble de nos personnels soignants et d'entretien, nos forces de sécurité intérieure, civiles et militaires,

La viticultrice que je suis a également une pensée particulière pour nos agriculteurs. À chacune et à chacun d'entre eux, je tiens à exprimer, au nom de mon groupe parlementaire, toute notre admiration et notre gratitude. J'exhorte chacun à remplir son devoir et à poursuivre le combat, où qu'il se trouve, quel que soit son rôle. Alors, la France pourra être fière de ses enfants et sera une nouvelle fois au rendez-vous de l'histoire.

Notre République, solidaire et fraternelle, démontre une fois encore qu'elle est debout lorsque l'essentiel est en jeu. Monsieur le ministre de l'intérieur, pouvez-vous indiquer aux élus de la République ce que le Gouvernement attend d'eux précisément ? Avec quels moyens, notamment techniques,

celles et ceux qui, demain, seront les acteurs de la protection de la nation française.

Devant cette asphyxie délibérée de l'hôpital, la casse de la santé et du secteur médico-social, la mobilisation du personnel n'a pas faibli. Depuis plus d'un an, il est en grève,

nous devons aborder les questions liées à cette épidémie dans un esprit de responsabilité. Rien n'est plus remarquable que l'attitude de nos soignants qui, en dépit d'un danger possible,

expression. Y aura-t-il assez de respirateurs, de brancards, de médecins, d'infirmières ? Combien de lits de réanimation sont-ils aujourd'hui ouverts ? Combien le seront dans les prochaines semaines ? D'autres hôpitaux de campagne sont-ils prévus dans notre pays ?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

Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, la France fait face à sa plus grave épidémie depuis un siècle.

8 700 morts, une propagation rapide de pays en pays, une mortalité qui touche sans choisir, mais d'abord les plus âgés et les plus vulnérables, des prévisions épidémiologiques alarmantes qui peuvent faire craindre, si la riposte était défaillante, des centaines de milliers de décès à travers le monde. La France est frappée de plein fouet et fait face avec détermination depuis janvier. Elle a recensé plus de 9 000 malades et déplore 264 morts à ce jour, un chiffre élevé et qui va s'accroître. Ni le Sénat ni l'Assemblée nationale ne sont épargnés, et je voudrais, monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, présenter mes voeux de très rapide et très complet rétablissement aux parlementaires, fonctionnaires et collaborateurs des assemblées malheureusement atteints. Cette crise sanitaire a également des répercussions majeures sur tous les aspects de la vie de la Nation. En quelques jours, nos modes de vie, nos priorités, nos habitudes, nos plaisirs les plus simples, nos préoccupations ont basculé. La vie économique, sociale et culturelle quotidienne s'est comme figée. Le Président de la République l'a dit, c'est une forme de guerre que nous menons. J'ai été personnellement frappé d'entendre la chancelière allemande, Mme Merkel, estimer hier qu'il s'agissait de la crise la plus grave que traversait l'Allemagne depuis 1945. Je m'inscris pleinement dans ces analyses : la période dans laquelle nous sommes entrés n'a rien de commun avec les crises économiques ou financières que nous avons connues depuis 1945. Elle aura des répercussions dans nos vies individuelles et dans la vie de notre Nation, dont nul ne peut aujourd'hui mesurer l'intensité, mais dont nous sentons tous qu'elles seront majeures. Notre réaction, notre politique, notre stratégie peuvent être résumées par deux mots simples : faire face.

méticuleux et assez remarquable d'identification des cas contacts réalisé par les équipes médicales du ministère de la santé et les responsables locaux. Notre stratégie n'a pas varié : empêcher aussi longtemps que possible le virus de s'installer et en freiner au maximum la progression.

Les enfants semblent épargnés, mais la gravité augmente avec l'âge et les autres fragilités sanitaires, avec une mortalité importante pour nos anciens.

et ensuite de ralentir la progression du virus, de façon à aplatir le pic épidémique. C'est ce qui nous permettra de diminuer considérablement le nombre d'urgences qui affluent chaque jour Nous limiterons ainsi le risque d'asphyxie de nos services de réanimation et nous leur donnerons le temps de s'organiser. Nous donnerons aussi le temps aux producteurs de masques, de solutions hydroalcooliques et de respirateurs de fournir les équipements dont nous avons besoin. En freinant la progression de la maladie dans la population, nous nous rapprochons également du moment où, nous l'espérons, nous disposerons de traitements, voire de vaccins. Dans certaines régions, en particulier dans l'Est et en Île-de-France, les hôpitaux font face à un afflux massif de patients nécessitant des soins urgents. Malgré la très forte pression qui s'exerce sur lui, notre système de soins tient le choc, avec bien sûr des différences d'intensité entre les territoires et au prix d'efforts considérables. Nous le devons aux capacités d'anticipation et d'organisation des personnels soignants, que nous tenons tous à citer, car ils sont en première ligne dans cette bataille : les médecins, les internes, les infirmiers, les aides-soignants, les médecins retraités, les étudiants.

Je veux leur redire ici notre reconnaissance, celle de la République, la nôtre, celle de millions de Français qui l'expriment parfois avec des mots, des actes ou des gestes qui ont frappé l'imagination de nos concitoyens. Je veux les assurer de notre totale mobilisation pour qu'ils puissent disposer, dans les meilleures conditions, des moyens dont ils ont besoin. Notre stratégie comporte aussi une dimension européenne et internationale. Dans le monde ouvert où nous vivons, rien ne peut être accompli sans coopération internationale, mais il est de fait que nous sommes confrontés à un défi inédit. Nous avons immédiatement saisi les institutions de l'Union européenne de la nécessité de coordonner nos réponses. Ce n'est pas un secret : quand, à la demande pressante de la France, les ministres de l'intérieur, d'une part, et les ministres de la santé, d'autre part, se sont réunis en février, beaucoup estimaient qu'il n'y avait pas lieu de le faire.

et la réalité que nous connaissons aujourd'hui. C'est en grande partie grâce à l'insistance du Président de la République et du Gouvernement que des mesures de coordination minimales ont pu être prises aux frontières comme en matière de politique sanitaire. Il est clair que la responsabilité première incombe aux États, mais nous devons pouvoir compter sur les avis de l'OMS, partager nos réponses, mieux coordonner les efforts de recherche de traitements et de vaccins. C'était l'objet du sommet exceptionnel des 7 et 16 mars derniers. C'est aussi par la solidarité européenne et internationale que nous pourrons aborder les dramatiques conséquences économiques de la crise. Je salue à cet égard les récentes décisions de la Banque centrale européenne. La bataille sera longue, et nous savons que le bilan en sera lourd. Nous agissons terriblement contraints par le temps,

de traitement, même si -rayon d'espoir -des essais cliniques et des tests, autorisés d'ailleurs avec une célérité jamais vue dès le mois de février, laissent espérer des découvertes en la matière. Nous agissons dans des délais très courts, selon quelques principes simples que je voudrais résumer. L'humilité, d'abord : elle oblige à reconnaître que l'on ne sait pas tout, l'on peut se tromper et que l'on doit, dans ce cas, corriger sans délai la trajectoire sans s'obstiner, que l'on doit s'inspirer aussi de ce que font les autres pays ayant le redoutable privilège de nous précéder parfois d'une semaine ou de quelques jours sur la courbe épidémique.

questions. Leurs avis sont souvent traversés d'opinions, d'analyses différentes, et le consensus scientifique n'est

Toutes nos décisions politiques prennent appui sur ce que les scientifiques peuvent nous indiquer dans l'océan d'incertitudes dans lequel nous nous trouvons. Dernier principe, la transparence à l'égard des Français.

il y aura, c'est bien légitime, des discussions, des contestations et des polémiques sur nos choix. Les discussions, les contestations, même rugueuses, sont bienvenues : elles nous font avancer, nous en avons besoin.

Mais les polémiques, que je classe dans une autre catégorie, peuvent nous distraire, nous retarder. Mesdames, messieurs les sénateurs, mon objectif est de conserver toute mon énergie pour avancer. Ce dont je veux vous assurer, c'est que le Président de la République, le Gouvernement et moi-même sommes engagés sans réserve, avec l'humilité que commande le moment, mais avec une détermination absolue, et décidés à assumer les choix que dictent notre compréhension de la situation, nos forces, nos vulnérabilités, sur la base des recommandations du corps médical. Je tiens à vous remercier, monsieur le président, ainsi que le président de l'Assemblée nationale, les présidents de groupe parlementaire, les présidents de commission

Je salue également l'esprit républicain dans lequel les formations politiques se sont inscrites. Devant le Sénat, je tiens à rendre hommage à tous les élus locaux, à tous les fonctionnaires nationaux, régionaux, départementaux, municipaux, qui donnent sans compter leur temps et leurs efforts. L'évolution rapide de l'épidémie nous a conduits, en fin de semaine dernière, à donner, sur la recommandation des médecins, un nouveau coup de frein et à décider, lundi, le confinement des populations sur le territoire national. Ces mesures sont massives, draconiennes ; jamais notre pays n'avait connu des mesures de restriction aussi générales et rigoureuses sur l'ensemble de son territoire. J'ai parfaitement conscience de l'effort qu'elles représentent pour des millions de Français. ils doivent à la fois s'acquitter de leurs obligations professionnelles, fût-ce à distance, continuer à gérer les contraintes familiales, les engagements de toutes sortes qu'ils ont pu souscrire,

-que ces mesures sont indispensables, qu'elles sont les seules efficaces pour soulager nos soignants et protéger ceux que nous aimons, que la négligence, la légèreté, l'insouciance que l'on constate parfois encore dans nos rues sont- je pèse mes je pèse mes mots -irresponsables et doivent laisser place à une prise de conscience totale de la responsabilité de chacune et de chacun d'entre nous dans le combat que nous avons engagé. L'épidémie et ces mesures de restriction ont, vous le savez, des répercussions d'une extrême gravité sur notre économie. Dans de nombreux secteurs- je pense au transport aérien, à l'hébergement, aux activités culturelles et sportives, à l'événementiel, à la restauration, au commerce de détail non alimentaire -, les chutes de chiffre d'affaires sont proches de 50 %, voire de 100 %. Cette crise bouleverse aussi l'ensemble de nos relations économiques, juridiques, administratives, ainsi que le fonctionnement de nos institutions démocratiques, nationales et locales. Lors de ses deux adresses aux Français, le Président de la République a annoncé des mesures massives pour contrer l'épidémie, pour soutenir financièrement les personnes les plus fragiles, les salariés, les indépendants, ainsi que les entreprises, grandes et petites. Ces mesures sont attendues, elles sont nécessaires, d'abord pour que les Français puissent se concentrer sur le seul objectif qui vaille : protéger leur santé, celle de leurs proches, celle de leurs concitoyens. Elles sont aussi nécessaires pour ne pas ajouter de l'angoisse sociale, économique, à l'angoisse que suscite déjà l'épidémie. Elles sont nécessaires pour que la vie économique et sociale de notre pays puisse reprendre le plus vite possible une fois la crise sanitaire derrière nous. Tout l'enjeu consiste maintenant à traduire ces mesures dans notre législation pour qu'elles puissent produire produire leurs effets dans le délai le plus court possible. L'urgence commande, et le Parlement est appelé à les discuter et à les voter aussi vite que possible, mais l'urgence ne saurait aller sans respect de l'indispensable pouvoir de contrôle des deux assemblées. C'est cet équilibre entre la rapidité de la décision dans la bataille et l'impératif absolu du contrôle démocratique que nous nous sommes employés collectivement à respecter. C'est ainsi que j'ai l'honneur de vous présenter les projets de loi adoptés hier en conseil des ministres : un projet de loi d'urgence, assorti d'un très court projet de loi organique, ainsi qu'un projet de loi de finances rectificative. L'ensemble de leurs dispositions visent à atteindre quatre objectifs. Le premier, c'est de protéger à tout prix, quoi qu'il en coûte, la population contre l'épidémie. Le deuxième objectif consiste à prendre les mesures économiques et sociales exceptionnelles que la situation impose. Le troisième objectif est d'adapter très temporairement nos règles de droit aux bouleversements que nous connaissons dans nos relations économiques ou administratives, que l'on soit une entreprise ou un particulier. Ces dispositions visent enfin, quatrièmement, à tirer les conséquences de l'impossibilité que nous avons constatée d'organiser le second tour des élections municipales ce dimanche.

Ce report, nous l'avons décidé lundi après avoir consulté le conseil scientifique et les forces politiques, parce que l'accélération de la propagation du virus le rendait indispensable. Je souhaite revenir sur cette question qui suscite, et c'est bien normal, discussions et interrogations.

et, nous le savons, seules des circonstances absolument exceptionnelles peuvent permettre d'en modifier le calendrier, sur la base, dans toute la mesure du possible, du consensus des forces politiques. Dès le mois de février, lorsque j'ai réuni à Matignon les partis et les groupes politiques pour les informer précisément de la situation sanitaire, la question du maintien du scrutin municipal a été abordée. À l'époque, sur l'avis unanime des autorités scientifiques, nous avons considéré que ce scrutin pouvait et devait être maintenu. À partir de ce moment, nous avons systématiquement interrogé les spécialistes sur les conditions d'une organisation sûre de ce scrutin Leur réponse a été de recommander la sensibilisation de nos concitoyens et de tous ceux qui allaient procéder ou faire procéder aux opérations électorales à ces consignes de sécurité et à ces gestes barrières grâce auxquels les contaminations pouvaient être évitées. Il n'y avait donc, à leurs yeux, pas de risque plus élevé à voter qu'à procéder à des actes courants de la vie quotidienne, comme faire les courses ou emprunter les transports en commun. Jeudi dernier, avant le premier tour, alors que nous décidions des premières mesures lourdes de confinement, la question du report a de nouveau été examinée.

consultés, parfois informellement, c'est vrai, nous ont dit que, sur la base des informations dont ils disposaient, ils considéraient que les opérations électorales, pour autant qu'elles soient bien organisées, que les consignes de sécurité soient bien mises en oeuvre et respectées, pouvaient se tenir, et le conseil scientifique a confirmé son analyse précédente. Samedi, enfin, veille du vote, alors que nous resserrions encore les mesures de confinement, nous avons de nouveau consulté les experts, qui ont confirmé leurs recommandations. Qu'aurait-on dit, mesdames, messieurs les sénateurs, si, par un décret pris nuitamment

Lundi, nous avons donc décidé, après une nouvelle consultation des forces politiques, le report du second tour, que recommandaient les experts du conseil scientifique. Il faut maintenant tirer les conséquences de cette situation sur notre vie municipale. Les solutions que préconise le Gouvernement, qui trouvent leur traduction dans le projet de loi qui vous est présenté, reposent sur deux principes. dans toutes les communes où le premier tour n'a pas permis d'élire l'ensemble du conseil municipal, le texte fixe la tenue du second tour au mois de juin, sous réserve bien sûr que nous ayons alors contenu l'épidémie. Pour nous en assurer, et pour anticiper, le Gouvernement remettra un rapport au Parlement au milieu du mois de mai 2020. Ce rapport se fondera sur les observations du conseil scientifique.

ce rapport indiquera s'il est possible d'installer les conseils municipaux dans les communes où le premier tour a permis d'élire l'ensemble du conseil.

Cette solution que nous proposons se fonde, d'une part, sur l'avis du président du conseil scientifique, qui, consulté aujourd'hui, a indiqué que les conditions sanitaires pour l'installation des conseils municipaux, prévue par le code électoral entre demain matin et dimanche, n'étaient plus réunies, et, d'autre part- j'exprime ici ma reconnaissance au président du Sénat, à l'ensemble des présidents de groupe et au président de la commission des lois sur une analyse partagée des contraintes qui pèsent sur nous. Cette analyse a permis de construire une solution qui m'apparaît à la fois simple, claire et raisonnable. Elle implique la prorogation des mandats des sortants, afin d'assurer la continuité de l'administration des affaires locales. Elle impose au Gouvernement d'expliquer ses choix au Parlement à une date fixée par le projet de loi au 10 mai. Par ailleurs, le projet de loi prévoit également des règles spécifiques pour clarifier un certain nombre de cas. Je pense à celui des communes de moins de 1 000 habitants, dans lesquelles il arrive que des candidats soient élus au premier tour sans que le conseil municipal soit au complet. de loi prévoit aussi des règles relatives au bon fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale. Sur tous ces points, nous sommes évidemment ouverts à des améliorations, avec toujours pour objectif de recueillir le consensus le plus large possible. Le titre II prévoit

à prendre, « en cas de menace d'épidémie », toute mesure pour protéger la santé de la population. C'est sur ce fondement légal que nous avons pris les mesures que la propagation de l'épidémie imposait.

méritaient un cadre plus respectueux de notre vie démocratique qu'un simple arrêté ministériel. Il s'agit non pas de choisir entre protection de la santé publique et démocratie, mais de protéger la santé de nos concitoyens, face à l'urgence, tout en respectant pleinement le rôle du Parlement et les garanties fondamentales.

Il prévoit une déclaration par la voie d'un décret en conseil des ministres, dont la prorogation au-delà d'un mois devra être autorisée par la loi. Dans une démocratie, on ne peut pas gérer l'exception sans le Parlement ; on ne peut pas déroger aux libertés aux libertés essentielles sans en appeler à son contrôle. Le cadre que nous proposons est objectivement plus satisfaisant et plus respectueux du Parlement que celui qui prévaut à ce jour. La comparaison entre les deux régimes d'état d'urgence s'arrête là. Il s'agit évidemment non pas d'autoriser des perquisitions, des assignations à résidence, mais de prendre des mesures générales de protection de la population. Pour bien en marquer la nature sanitaire, nous avons décidé de faire figurer ce dispositif dans le code de la santé publique. Les mesures envisagées auront donc toujours un objectif sanitaire et leur proportionnalité sera évidemment contrôlée. ne me demandez pas d'en dresser à l'avance la liste : l'expérience des dernières semaines nous appelle à l'humilité en la matière. Veillons aussi, ensemble, à ce que la loi nous permette de nous adapter si l'épidémie devait sévir par pics successifs ou selon des formes variées sur les territoires. Je l'ai dit, la situation actuelle est sans précédent ; jamais la vie ne s'était arrêtée à ce point dans notre pays. À bien des égards, nous évoluons dans une forme d'inconnu. Nous avons pu anticiper un certain nombre de conséquences de cette vie en quelque sorte soudainement mise sous cloche. Dans d'autres domaines, nous ne connaissons pas avec certitude la nature, la durée et l'étendue des mesures que nous aurons à prendre pour nous adapter. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande au Parlement, au travers du titre III du projet de loi d'urgence, de l'habiliter à prendre de nombreuses mesures par ordonnances. Ces mesures visent d'abord à mettre en oeuvre les décisions que le Président de la République a prises pour protéger les Français. Je pense par exemple aux mesures économiques de soutien à la trésorerie des entreprises, aux aides directes, à l'assouplissement des règles commerciales et de procédure civile ou aux délais que nous voulons accorder aux très petites entreprises pour payer leurs factures d'eau ou d'électricité. Bien souvent, ce sont des mesures de survie pour nos restaurateurs, nos artisans, nos commerçants. Ces mesures sont aussi destinées à assouplir l'organisation du travail, à faciliter, le cas échéant, le recours aux congés payés, à la formation, et à indemniser, à des niveaux bien plus élevés qu'aujourd'hui, le chômage partiel, de manière à éviter des licenciements massifs, qui seraient catastrophiques sur les plans social et économique. Ces mesures vont également permettre à des millions de foyers de ne pas souffrir de pertes brutales de revenus, comme cela pourrait être le cas dans d'autres pays. Ces mesures d'exception visent en outre à faciliter la garde des enfants, alors que nous avons décidé de fermer, toujours pour freiner l'épidémie et la circulation du virus, les structures d'accueil de jeunes enfants. Ces mesures, enfin, ont vocation à protéger les plus fragiles. Nous mettons ainsi en oeuvre les engagements du Président de la République en suspendant les expulsions locatives ou en prenant des dispositions exceptionnelles en faveur des personnes qui souffrent d'un handicap. Nous leur devons évidemment notre protection. Par ailleurs, nous avons maintenu ouvertes toutes les places d'hébergement d'urgence et mis en place des dispositifs d'accueil des personnes à la rue. À côté de ces mesures de soutien, le projet de loi vise à autoriser le Gouvernement à prendre des dispositions de bon sens.

Ces mesures de bon sens visent également à adapter les délais légaux et les procédures dans les juridictions civiles, pénales ou commerciales, afin de garantir les droits des citoyens. En d'autres termes, pas un Français ne doit perdre un droit ou prendre un risque inutile pour sa santé à cause de règles de droit qui se justifient parfaitement dans des conditions normales, mais qui se révéleraient hors de propos dans un pays confiné. Toutes les dispositions que nous suspendons s'appliqueront de nouveau à la fin de la période d'épidémie, mais ces mesures d'assouplissement, de soutien ou de suspension doivent nous aider à passer le gros de la tempête, avant que la situation ne redevienne à peu près normale. Cette crise sanitaire grave, terrible même, nous la surmonterons. Ensuite, la vie économique, sociale, politique reprendra, le plus vite possible. on le sait, aura des conséquences graves sur l'activité économique dans notre pays. Tout l'enjeu est d'aider nos entreprises et leurs salariés à franchir ce cap. Dans cette perspective, le Président de la République a fixé un objectif clair : nous devons soutenir nos entreprises et nos emplois quoi qu'il en coûte.

Nous consacrerons également, avec les régions, dont je tiens à saluer ici l'engagement, près de 1 milliard d'euros au fonds d'indemnisation dont bénéficieront les indépendants. Nous avons en outre prévu une provision de 2 milliards d'euros pour soutenir l'hôpital et faire face aux dépenses d'indemnités journalières. Le projet de loi de finances rectificative met par ailleurs en place un dispositif exceptionnel de garantie publique des crédits bancaires aux entreprises, à hauteur de 300 milliards d'euros, soit un montant comparable à ceux que les Allemands ou les Britanniques sont en train de mobiliser. Concrètement, il s'agit de faire en sorte que les banques continuent de prêter aux entreprises et de soutenir leur trésorerie. Les entreprises s'adresseront directement à leur banque et bénéficieront automatiquement d'un différé d'un an avant de rembourser leur prêt, qui pourra représenter jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires constaté en 2019. est massif et inédit. Il est, je le crois, à la mesure de la crise que nous connaissons, des risques que cette crise sanitaire fait courir à l'ensemble de notre économie. Comme vous le savez, le temps presse. Chaque jour, chaque semaine qui passe, ce sont des milliers d'entreprises qui se fragilisent, c'est la précarité qui menace. C'est la raison pour laquelle nous n'avons eu d'autre choix que de proposer au Parlement un examen de ces projets de loi dans des délais très contraints. Je remercie une nouvelle fois ses membres et les groupes des deux assemblées de leur volonté de s'accorder très vite sur les termes de ces textes et de faire prévaloir l'union. C'est dans le même esprit, selon la même volonté d'union nationale, que le Président de la République a demandé au Gouvernement de suspendre l'examen et la mise en oeuvre du système universel de retraite et l'application de certaines dispositions de la réforme de l'assurance chômage. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous savons tous que l'heure est particulièrement grave. La France affronte une grande épreuve ; elle combat un ennemi silencieux, invisible, aveugle. Dans le passé, nombreux ont été les scientifiques, les responsables politiques à redouter la survenue d'une crise sanitaire de cette ampleur. La vie a décidé qu'il reviendrait à ce ce Parlement, de l'affronter, aux côtés de nos 65 millions de compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Nous devons le faire dans l'unité, le calme, la discipline, le sang-froid, avec l'esprit de responsabilité et de fermeté qui a animé nos prédécesseurs dans des circonstances exceptionnelles. Cette bataille aura, je le sais bien, et on le voit déjà, sa part d'ombre avec ces vols, ces trafics, ces accapareurs et ces profiteurs, ces violences, cette légèreté, ces basses polémiques, parfois, qui ne sont que le triste reflet de ce que l'homme peut faire lorsqu'il est angoissé, lorsqu'il a peur ou lorsqu'il oublie qu'il fait partie d'une grande Nation. Mais elle connaîtra ses héros. Je les ai salués déjà, et je n'ai aucun doute que, dans la durée, d'autres se révéleront. Elle connaîtra ses victimes, aussi, et nous devons en limiter le nombre. Elle connaîtra ses soldats du quotidien, toutes celles et tous ceux qui s'appliqueront avec discipline, avec acharnement, avec inventivité, avec fraternité à respecter les règles tout en maintenant l'espoir, le sourire et la vie. Nous sommes, mesdames, messieurs les sénateurs, une grande Nation, et si les facilités des temps tranquilles nous le font oublier parfois, au coeur de l'âme française, cette force, cette cohésion, cette grandeur qui me donnent une absolue confiance dans l'issue. Nous vaincrons ce virus avec nos forces politiques, économiques, scientifiques, culturelles, spirituelles aussi, avec tous les pays, toutes les communautés qui se liguent contre lui, et nous devrons être prêts, ensuite, à repartir d'un pied nouveau,

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, depuis les mesures drastiques prises par le Gouvernement il y a quelques jours, quelques semaines pour certaines d'entre elles, c'est la première fois que nous sommes réunis en séance publique. Le Gouvernement agit ; il appartient au Parlement de répondre présent pour contribuer à relever ce défi exceptionnel qui est lancé à notre pays

des difficultés auxquelles nous sommes collectivement confrontés. Cette voix des Français que nous portons, c'est aujourd'hui celle de l'inquiétude, de l'angoisse

et pour affronter les difficultés de l'épreuve que nous avons commencé à traverser et dont nous savons bien, hélas, qu'elle va s'aggraver au fil des prochains jours, avant

nous font un devoir plus grand encore que dans les temps ordinaires de jouer notre rôle constitutionnel et de ne pas laisser l'exécutif seul face à la crise, en prenant notre

pour arrêter des mesures exceptionnelles que, dans une grande démocratie, le Gouvernement ne peut assumer seul, mais que nous sommes prêts à lui permettre de prendre ou de consolider quand elles ont déjà été prises sur un fondement légal, dont vous avez souligné à l'instant qu'il n'était pas suffisant, ce qui justifiait donc que nous nous réunissions pour déterminer de nouvelles mesures législatives. Nous porterons pendant toute cette période l'exigence de dialogue dialogue et de transparence, autant que celle, impérieuse, d'unité nationale, parce que nous le devons à nos compatriotes.

de nos compatriotes. Chacun doit pouvoir dire : « Le virus ne passera pas par moi, parce que je fais ce qu'il faut faire pour l'éviter et contribuer ainsi à ce que la santé publique soit sauvegardée malgré la gravité de cette épidémie. » Je veux saluer ici l'esprit de discipline et de responsabilité qui prévaut aujourd'hui parmi les Français, après qu'ils eurent pris le temps d'intégrer la gravité de la situation et la menace qui pèse sur chacune et chacun d'entre nous.

est la disposition d'esprit dans laquelle la commission des lois a examiné le texte du Gouvernement. Elle a veillé à mettre au premier rang de ses préoccupations la sécurité sanitaire de nos concitoyens, pour contribuer à lutter le plus efficacement possible contre cette épidémie du Covid-19. Elle a donc veillé à ce que les autorités disposent des moyens d'action exceptionnels dont elles ont besoin pour faire face à la crise, pour prévenir les contaminations et pour assurer dans les meilleures conditions possible la prise en charge des malades. Elle s'est aussi attachée, dans ses travaux, à ce que les moyens mis en oeuvre, parfaitement dérogatoires dans notre État de droit, soient strictement proportionnés aux objectifs de sécurité sanitaire des pouvoirs publics, dont nous soutenons l'action de lutte contre ce fléau, en faisant en sorte que les restrictions apportées à l'exercice de libertés fondamentales ne soient que des restrictions strictement indispensables, pour une durée limitée et sous un contrôle renforcé du Parlement. Vous verrez, au moment de l'examen des articles, quelles conséquences nous en avons tirées. À ce stade de nos débats, je veux surtout insister sur la philosophie qui nous a inspirés. L'état d'urgence sanitaire permettra au Gouvernement de prendre par décrets des mesures restrictives. Nous voulons qu'elles soient limitées et qu'elles relèvent de catégories énoncées par le législateur. Les conseils municipaux et communautaires n'auront pas à être réunis pendant la période de confinement si les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas réunies. Les présidents de conseil communautaire resteront en place pour qu'il ne soit pas nécessaire de convoquer des réunions qui pourraient comporter plus de 200 participants dans certains cas. Les règles de quorum

Nous avons également fait en sorte que l'on s'écarte le moins possible des règles de droit commun. C'est pourquoi, pour la préparation du second tour des élections municipales, nous avons tenu à ce que les déclarations de candidatures soient déposées dans les plus brefs délais, afin d'éviter d'interminables négociations. Enfin, je veux saluer l'effort fait par le Gouvernement pour l'élection des maires et de leurs adjoints, prévue initialement vendredi, samedi et dimanche de cette semaine. Monsieur le ministre de l'intérieur, nous nous en étions entretenus dès hier soir avec Mme Braun-Pivet, mon homologue la présidente de la commission des lois de l'Assemblée nationale. Nous étions convenus que, si ces élections étaient maintenues, il fallait à tout le moins que des dispositions exceptionnelles soient prises pour que les conseils municipaux soient en mesure d'élire les maires sans que tout le monde soit présent, grâce à un assouplissement du régime des procurations et des règles de quorum. La discussion s'est prolongée.

sont les référents de nos concitoyens. Ils ont, parmi leurs attributions, des responsabilités en matière d'hygiène publique. Il est important que notre démocratie ne soit pas mise en suspens. Gageons au contraire que c'est grâce aux méthodes qui sont propres à notre démocratie que nous serons les plus forts, puisque tout le monde doit s'engager dans le combat pour maîtriser la grave situation d'épidémie que nous avons à surmonter.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, à intervalles réguliers dans son histoire, le peuple français a été menacé par des défis très graves. Il a toujours su se relever. Aujourd'hui, un tsunami sanitaire et économique a débuté, et la France, de nouveau, doit rester debout. La crise rappelle, à ceux qui l'auraient oubliée, la valeur inestimable de la solidarité nationale, de notre service public, et la formidable énergie collective qui anime notre Nation. Sachons rendre hommage à ces femmes et ces hommes qui oeuvrent, chaque jour, pour endiguer la crise ou en atténuer les effets. À la place qui est la mienne, je pense également à nos agriculteurs, à nos industriels, aux salariés du commerce, qui garantissent aux Français une alimentation suffisante, même quand les rayons des magasins sont assaillis par des consommateurs inquiets. Le choc économique actuel agit à la fois sur la demande et sur l'offre. Il affectera fortement notre modèle économique. Conjoncturellement, la France affrontera cette année une récession, peut-être pire que celle annoncée à ce stade par le Gouvernement, si la pandémie venait à durer.

Pouvez-vous nous confirmer que tous les professionnels sont visés par l'article 7, indépendamment de leur statut juridique, c'est-à-dire y compris les associations de l'économie sociale et solidaire ou les professions libérales, Vous évoquez un seuil de 70 % de perte de chiffre d'affaires pour le mois de mars, par rapport à mars 2019, pour être éligible au fonds de solidarité. Ce seuil nous paraît soit trop élevé,

La crise atteindra également structurellement notre modèle économique. Cette crise nous montre que nous sommes entrés dans une période de graves incertitudes géopolitiques, écologiques, sanitaires et donc économiques. Après les Trente Glorieuses, nous sommes sans doute entrés dans les « trente dangereuses des chocs qui mettent en cause notre modèle de société. Dans ce monde incertain, la France ne manque pas d'atouts, mais elle doit rester guidée par trois valeurs qui ont toujours fait corps avec le modèle français : la souveraineté, la responsabilité et la résilience. La souveraineté, tout d'abord, économique, numérique, énergétique ou alimentaire. La crise a montré, et la gaulliste que je suis en est convaincue, que nous devons cesser de croire aveuglément que nous pouvons compter sur les autres autant que sur nous-mêmes. Ne prenons pas à la légère notre destin économique ou alimentaire. À l'heure où nous importons une part significative de notre alimentation, nous devons nous interroger. La responsabilité, ensuite. L'État comme les collectivités territoriales auront une responsabilité immense. Ils devront réintroduire la notion de long terme et en finir avec un court-termisme qui nous désoriente. Qu'attendons-nous, monsieur le Premier ministre, pour suspendre les cotations boursières, Chacun, citoyen, consommateur, salarié, entrepreneur, devra modifier ses attitudes pour prendre en compte les conséquences collectives de ses décisions individuelles. La résilience, enfin. La France de demain doit repenser sa capacité à réagir aux défis. Le rôle de l'État doit évoluer : il sera plus régulateur, plus stratège. Il devra être plus économe en période de croissance, pour disposer de plus de ressources budgétaires en cas de crise. Le secteur privé doit réinventer de nouveaux modèles, de nouveaux services, en particulier dans le domaine numérique. Enfin, la société elle-même doit organiser sa propre capacité de résistance, une résistance sociale, générationnelle et solidaire. Résilience, souveraineté, responsabilité : voilà le cap qu'il nous faut fixer dans cette tempête ! Nous relèverons ce défi, monsieur le Premier ministre. La France et son peuple sont puissants

s'annoncent. La parole est à M. le rapporteur pour avis de la commission des affaires sociales. Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, les circonstances exceptionnelles qui nous réunissent aujourd'hui appellent des mesures exceptionnelles. Parmi les dispositions contenues dans le projet de loi ordinaire soumis à notre examen, la commission des affaires sociales s'est saisie pour avis du titre II, qui porte sur la création d'un état d'urgence sanitaire, ainsi que de l'article 7, qui prévoit l'habilitation du Gouvernement à prendre par ordonnances plusieurs mesures touchant au droit du travail ainsi qu'en matière sociale. Deux principes ont guidé notre examen de ce texte destiné à adapter notre droit à des circonstances exceptionnelles la nécessité et la proportionnalité, avec le souci de ne pas aller plus loin que ce que prescrit la situation difficile que nous vivons et que nous allons vivre encore pendant une période indéterminée, laquelle sera de toute façon très longue. le prisme de ces deux principes, il a semblé à la commission des affaires sociales que les dispositions de l'article 7 étaient nécessaires et proportionnées, à deux exceptions près. le titre II, en revanche, il est légitimement permis de s'interroger sur la nécessité d'un nouveau dispositif s'ajoutant au droit actuel. La création d'un état d'urgence sanitaire a répondu à la nécessité de conforter la base légale du décret pris par le Premier ministre le 16 mars dernier, dans lequel sont décrites les mesures de confinement, par définition restrictives de certaines libertés publiques, qui s'imposent à nous depuis bientôt trois jours. Le Conseil d'État a estimé indispensable la définition d'une nouvelle base légale, dont nous n'avons pas approuvé toutes les modalités. À notre sens, quatre difficultés pouvaient se présenter : premièrement, le caractère pérenne du dispositif proposé, qui s'ajoutait aux dispositifs existants en matière de mesures d'urgence sanitaire, au risque d'une concurrence juridique avec ces derniers ; deuxièmement, le périmètre initial des restrictions aux libertés d'aller et de venir ainsi que de réunion excédait très largement les mesures pour l'heure contenues dans le décret du 16 mars 2020 et faisait courir le risque d'une disproportion des mesures administratives troisièmement, certaines ambiguïtés relatives au rôle des différents acteurs ministériels, notamment s'agissant de l'articulation entre le ministre de la santé, revêtu d'une autorité hiérarchique d'exception sur les forces de l'ordre, et le ministre leur autorité naturelle, dont le décret du 16 mars continue de faire expressément mention ; quatrièmement, un élargissement des compétences du préfet, notamment lorsque ce dernier se trouve délégataire de l'ensemble des compétences normalement exercées par l'échelon ministériel. À l'ensemble de ces difficultés, nous estimons que les modifications introduites par la commission des lois apportent des corrections satisfaisantes, et la commission des affaires sociales s'en est remise à la nouvelle rédaction qu'elle propose pour l'état d'urgence sanitaire.

de l'urgence sanitaire, dont nous voyons aujourd'hui qu'il ne peut se satisfaire d'interventions législatives précipitées. Nous ne pourrons pas faire l'économie d'une réflexion approfondie. Ce ne sont certainement pas les conditions dans lesquelles nous légiférons aujourd'hui, sur le fondement d'un texte connu seulement dans la soirée d'hier, qui permettront d'élaborer un dispositif d'exception pérenne et proportionné. Sur l'article 7, je voudrais dire que les circonstances exceptionnelles ne doivent pas être vues comme l'occasion de recycler des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel. Je pense aux assistantes maternelles. Nous devons veiller en toutes circonstances à ne pas porter des atteintes démesurées aux droits des salariés. C'est le sens de l'amendement de la commission des affaires sociales sur le régime des congés payés. Enfin, la commission des affaires sociales a rappelé que la protection des salariés était une obligation de résultat pour l'employeur. Le défaut de protection suscite des angoisses légitimes et n'est pas acceptable s'agissant de personnes dont l'activité est essentielle à la vie du pays. Mes chers

souligne la gravité de la crise à laquelle notre pays est confronté, comme bien d'autres dans le monde. Notre présence aujourd'hui, dans un Paris confiné, souligne aussi la volonté du Parlement d'être là, de tenir son rang et de conserver à la République un équilibre des pouvoirs nécessaire en toutes circonstances. Oui, la France est en situation d'urgence, de grande urgence sanitaire. Le virus Covid-19 se répand ; l'épidémie gagne et des mesures extrêmes, lourdes sont bien entendu nécessaires pour endiguer le mal. Avant toute chose, je le dis à nos compatriotes : prenez soin de vous, restez chez vous, protégez les autres par votre prudence ; respectez les consignes d'hygiène, ces fameuses barrières ; faites grandir la solidarité, ce mot que que beaucoup réservaient à l'histoire ; soutenez ceux qui, vulnérables, souffrent particulièrement de cette situation ; bien entendu, affichez un soutien sans faille aux personnels de santé, qui, dans des conditions d'une difficulté inimaginable, affrontent la maladie. nous les applaudissons, celles et ceux qui, malgré un manque de moyens criant, malgré la disette imposée au monde de l'hôpital depuis des années, sont là, debout, jour et nuit, alignant les heures supplémentaires. Comment ne pas noter ici le rôle majeur joué par les femmes, à l'hôpital comme dans les Ehpad, ou encore dans les magasins d'alimentation, où elles sont en première ligne ? Oui, monsieur le Premier ministre, il y a urgence, grande urgence ! Notre groupe fera sien l'appel à l'unité de la Nation pour franchir cette épreuve dramatique. Aujourd'hui, comme en d'autres temps de l'histoire de notre pays, nous faisons preuve de responsabilité et ne souhaitons alimenter aucune controverse. Le temps viendra, mais l'urgence, c'est de sauver des vies concentrés sur les faits, sur les attentes, sur les besoins. Le projet de loi d'urgence présenté pour faire face à l'épidémie comporte des mesures nécessaires, comme celles relatives au confinement, mais il ne porte aucune rupture- mot pourtant mis en avant par Emmanuel Macron lui-même, jeudi dernier -avec les désastreuses politiques de santé publique de ces dernières années, qui nous ont amenés là où nous en sommes aujourd'hui. La situation de l'hôpital dénoncée tout à l'heure avec force par mon amie Laurence Cohen est d'une extrême gravité pour les personnels et les patients. Emmanuel Macron a pourtant affirmé, martelant son « quoi qu'il en coûte », que les moyens allaient être donnés à la santé, « qui n'a pas de prix », selon lui. « Ce que révèle cette crise », a-t-il noté, « c'est qu'il y a des biens et des services qui doivent être placés en dehors des lois du marché. Or rien n'est prévu à cette heure dans le projet de loi de finances rectificative. Or, « en même temps », ces textes sont encore et toujours marqués, encadrés, corsetés par la loi du marché. Comment ne pas voir que ce projet de loi d'urgence, en dehors des mesures d'ordre public et de soutien aux entreprises qu'il contient, fait peu de place à l'urgence sanitaire en elle-même, c'est-à-dire à une aide massive, immédiate, à la hauteur de l'état de crise que nous vivons ? Nous attendions par exemple des mesures pour accroître en urgence la production de masques, pour développer les tests, pour rendre plus efficace le confinement pour les personnels de santé, bien sûr, mais aussi pour celles et ceux qui sont en contact avec la population, comme les les policiers, les pompiers, et d'autres professions encore. Le soutien à l'économie, fondamental, occulte de manière un peu trop manifeste le soutien à notre système de santé. notre système de santé. Nous n'acceptons pas le poids que vous faites peser sur les salariés, encore et toujours première variable d'ajustement de la gestion des entreprises. Vous avez renoncé à l'interdiction des licenciements, pourtant annoncée par Mme Pénicaud lundi, et vous appelez les entreprises à la raison. Nous proposons, pour notre part, qu'aucune suppression d'emploi ne puisse avoir lieu durant cette période d'urgence. Vous remettez en cause, pour une durée indéfinie, le droit des salariés aux congés payés et aux RTT, ainsi que les 35 heures. Vous généralisez le travail du dimanche. Ces propositions sont

Ce projet de loi pose également un problème démocratique. Nous comprenons que la situation impose d'agir vite et de disposer d'une liberté d'action, mais le Parlement ne saurait être mis sur la touche en renvoyant à un, voire voire deux mois, un premier vote d'approbation de votre politique, alors qu'un délai de douze jours était prévu lors des états d'urgence précédents. De plus, l'introduction de cette nouvelle catégorie d'état d'urgence dans le code de la santé publique ne revient-elle pas à faciliter sa mise en oeuvre future ? C'est pourquoi nous proposons la mise en place d'un comité national de suivi de l'état d'urgence sanitaire pluraliste pour accompagner et contrôler l'action du Gouvernement. C'est une

monsieur le ministre de l'intérieur, d'avoir réuni cet après-midi les présidents de groupe pour échanger sur le report de l'élection des maires, prévue dès ce week-end, mais vous comprenez bien que l'on ne peut pas continuer à fonctionner ainsi, surtout si, malheureusement, cette crise sanitaire devait se poursuivre et s'aggraver encore. C'est pourquoi mon groupe insiste sur la création de ce comité de suivi pluraliste, qui devrait se réunir, selon nous, chaque semaine

Monsieur le Premier ministre, cette grave crise sanitaire qui traverse la planète pose des questions fondamentales à l'humanité. La mondialisation sauvage, cette mondialisation financière qui privilégie à outrance le profit sur l'humain, sur l'humain, ne pourra pas suivre son cours. Beaucoup pensaient que c'est le réchauffement climatique qui imposerait en premier lieu les changements et les ruptures inéluctables. Malheureusement, c'est un virus au coeur de l'homme, au coeur de l'humanité, qui peut ouvrir la conscience de ceux qui ne croient qu'à l'argent ... Nous ne nous opposerons pas à ce texte, mais, pour l'heure, nous réservons notre vote final. monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, jamais un réalisateur de films catastrophes n'aurait imaginé un tel scénario. Au début de l'hiver, sur les étals d'un marché chinois, où l'on vend pêle-mêle champignons et plantes médicinales improbables, animaux à plumes et à poils, morts et vivants, où des chauves-souris nichent dans les trous des plafonds, un vieil homme achète à la découpe un morceau de l'animal le plus bizarre au monde, qui ressemble à un rat entièrement couvert d'écailles. Il l'emporte chez lui, le prépare, le mange et meurt en quelques jours, bientôt suivi par d'autres clients du même marché. Les médecins signalent l'affaire aux autorités. Les apparatchiks locaux, terrifiés à l'idée, assez plausible en Chine, d'être châtiés pour un événement dont ils ne sont pas responsables, menacent les soignants des pires sanctions s'ils l'ébruitent. Un jeune médecin passe outre ; son compte WeChat est bloqué, mais son post a commencé à circuler. Il meurt quelques jours plus tard de la maladie qu'il vient de découvrir. Entre le 17 novembre, date de l'apparition du premier cas, et l'annonce en janvier par les autorités chinoises de l'émergence d'un nouveau virus, deux mois se sont écoulés. Un petit foyer d'infection qui aurait pu être contenu va donner naissance à une pandémie. Ce n'est là que le début du film. La scène suivante se déroule dans un palais à Riyad. La Chine est à l'arrêt, le cours du pétrole vacille ; l'OPEP propose une réduction commune de la production à Poutine, qui refuse. Mohammed ben Salmane se venge en cassant les prix pour étouffer son concurrent : la guerre du pétrole entre l'Arabie saoudite et la Russie a commencé. À l'ouverture des marchés, le lundi 9 mars, les cours du Brent s'effondrent. Wall Street s'affole. La décision de l'Italie de confiner sa population fait comprendre le choc de demande qui va survenir. La dégringolade de la bourse se transforme en panique : le Vix, l'indice de la peur, s'envole. Les coupe-circuits des trois grands indices américains s'activent automatiquement. Les marchés européens plongent. Dernière séquence : une série de plans sur des dizaines d'écrans d'internautes. L'épidémie s'est transformée en « infodémie ». Les réseaux antisociaux affichent les chiffres les plus alarmistes, promeuvent les médecines farfelues, les bains d'eau chaude et les huiles essentielles. Les chaînes d'information, en concurrence effrénée, n'arrivent plus à trouver assez d'« experts ». À ceux de premier plan succèdent les deuxièmes et troisièmes couteaux, qui répètent en boucle ce qu'ils viennent de voir sur une chaîne concurrente ou disent n'importe quoi. Plus personne n'y comprend rien, la peur s'installe. Ce film, que même Orson Welles n'aurait osé imaginer, c'est l'état du monde aujourd'hui. Personne n'en connaît le dénouement. Face à cette crise mondiale, notre premier impératif est l'humilité. Nous sommes réunis pour décider des mesures qui vont s'imposer à notre pays. Jusqu'à présent, à quelques outrances près, l'union sacrée a prévalu. Si cet hémicycle, ou celui de l'Assemblée nationale, devait se transformer en une tribune politicienne, les Français ne nous le pardonneraient pas. Ils attendent des actes, et non des roulements de mécaniques. La question n'est pas de s'écharper sur l'opportunité d'avoir maintenu le premier tour des élections municipales ou sur la date de réunion des conseils municipaux. Prenons garde à ne pas être déclarés hors sujet.

il est essentiel de faire confiance aux autorités sanitaires et à leurs efforts quotidiens de transparence devant la marée des, du complotisme et de la peur. Il peut leur arriver, il leur est déjà arrivé de ne pas avoir toutes les réponses face à un ennemi inédit ; je suis en tout cas certain que les réponses qu'ils ont sont plus pertinentes que celles de leurs contradicteurs. contradicteurs. Il s'agit également, bien sûr, d'une crise économique et sociale. Elle sera tout aussi grave et pose un dilemme effrayant : prendre des mesures de confinement trop drastiques, c'est tuer l'économie ; ne pas en prendre, c'est laisser mourir des Français.

Cette crise, en quelques jours, a changé les Français. Jusqu'à dimanche dernier, les journaux du monde entier s'étonnaient de ce peuple incurable, rebelle à toute discipline, se réunissant par milliers dans les parcs sous le soleil.

Comme aux grands moments de leur histoire, ils se comportent en citoyens. Je vais me risquer à un pronostic : je ne suis pas pessimiste. Les exemples de la Chine- une fois les mensonges terminés -et de la Corée du Sud démontrent qu'avec des mesures adaptées la victoire sur l'épidémie est une question de semaines, et non de mois. C'est la voie que nous sommes en train d'emprunter. Quant à la crise économique, elle n'a rien à voir avec celle de 2008. Elle est beaucoup plus profonde, mais elle sera, je le crois, beaucoup plus courte. Lorsque la pandémie cessera, le monde entier sera saisi d'une frénésie de consommer, de voyager, d'aimer, en un mot de vivre- espérons-le d'une manière plus respectueuse de notre planète qu'aujourd'hui. Il n'y a rien qui s'oublie aussi vite que les guerres, les catastrophes ou les épidémies, une fois les beaux jours revenus. Je ne dis pas cela au hasard, mais pour l'avoir vécu, souvent, dans des pays bien plus vulnérables que le nôtre. C'est aussi ce que nous disent les livres d'histoire. Cette capacité d'oublier le malheur -peut-être faudrait-il dire « de le

République estime que nous sommes en guerre et assure que l'État soutiendra financièrement notre système de santé et notre économie, « quoi qu'il en coûte ». Rares sont les situations où l'urgence sanitaire est à ce point caractérisée. Le coronavirus a déjà infecté 200 000 personnes à travers le monde ; plus de 8 200 malades sont décédés. Le nombre de cas recensés en France est en constante augmentation. Désormais, l'Europe constitue le premier foyer de cette terrible pandémie. pourtant théoriquement suffisantes, n'ont pas été suivies par un grand nombre de nos concitoyens. Aussi le Gouvernement a-t-il dû renforcer les mesures de précaution. Cette situation sanitaire nous oblige à faire preuve de responsabilité, de réactivité, d'adaptation et de solidarité. Le présent projet de loi en est une illustration. Son titre II donne une base juridique spécifique à l'urgence sanitaire en répartissant les pouvoirs entre le Premier ministre, le ministre de la santé et, par délégation, le représentant de l'État. La durée de l'urgence reste encadrée et un comité scientifique est institué. Les temps à venir seront éprouvants pour nos professionnels de santé, qui savent toujours faire passer l'intérêt de leurs patients avant le leur. Toutefois, de nombreux témoignages inquiétants nous parviennent quant au manque de matériels pour nos soignants. Sans ces matériels, c'est la capacité de notre système de santé à combattre cette pandémie qui est mise en danger. C'est pourquoi je tiens à saluer les initiatives de certains industriels français, grands ou petits, qui produisent désormais des masques ou du gel hydroalcoolique, essentiels pour sécuriser l'activité des soignants, mais aussi celle des aides à domiciles, qui en ont grand besoin.

pour permettre à notre système de santé de réagir plus vite et d'être mieux préparé. Il faudra aussi que les réponses sanitaires soient coordonnées au moins à l'échelon européen, si ce n'est au niveau mondial. À la crise sanitaire sans précédent que vivent les Français s'ajoute une crise économique majeure dont les conséquences sont à la fois immédiates et de long terme immédiates, car la gradation des mesures de protection, jusqu'au confinement généralisé, empêche le fonctionnement d'une très large partie de notre économie ; de long terme, car cette paralysie aura des conséquences sur la pérennité des entreprises, sur l'emploi des salariés et sur notre modèle économique général. Afin de limiter les conséquences économiques pour les entreprises et de garantir le pouvoir d'achat des Français, le présent projet de loi prévoit un important train de mesures à prendre par voie d'ordonnances. Ces mesures correspondent aux annonces de l'exécutif. Le Gouvernement réagit de manière globale. Il me semble avoir pris la mesure des difficultés que rencontrent les entreprises, en particulier les TPE-PME et les artisans. Nous saluons les mesures présentées, en particulier celles qui visent à soutenir la trésorerie des entreprises, la mise en place d'un fonds de financement alimenté par l'État et les collectivités locales, mais aussi celles relatives au droit du travail, en particulier à l'indemnisation du chômage partiel. Toutefois, une interrogation persiste quant au report du versement des cotisations Urssaf pour les petites entreprises, voire à leur remboursement pour celles qui les auraient acquittées par avance. par avance. La question de l'arrêt des chantiers se pose, ainsi que celle du recours au dispositif d'activité partielle pour les entreprises concernées. Par ailleurs, nous aurions aimé savoir dans quelle mesure les assurances privées pourront être mobilisées au titre des garanties de pertes d'exploitation, par exemple pour les restaurateurs. Enfin, cette crise devra nous conduire à nous interroger sur nos orientations économiques et sur notre modèle de développement. Elle suscite une réflexion sur la relocalisation des activités économiques. Cela nécessitera d'accompagner les entreprises pour qu'elles fassent ces choix cruciaux, mais aussi, peut-être, de réinvestir dans la formation et l'apprentissage pour retrouver des compétences qui ont souvent été perdues du fait des délocalisations. Nous souhaiterions savoir si le Gouvernement réfléchit déjà à une forme de grand plan de relocalisation et de formation.

En entendant les Français applaudir à leurs fenêtres nos soignants, au front dans cette guerre contre l'épidémie, on sent que la démocratie repose non seulement sur une fraternité, mais aussi sur un sens civique, une vertu, une pratique morale.

de la notion de service public, qui fait partie de notre ADN républicain et n'est pas incompatible avec le développement du monde économique privé. Dans cette épreuve, la démocratie doit demeurer exigeante. Elle n'est pas plus faible qu'un régime autoritaire quand il faut affronter les périls sanitaires. Nous en ferons la preuve, en ne confondant jamais vitesse et précipitation. Surmontons la tension entre l'autorité du Gouvernement et la continuité démocratique exprimée dans le contrôle parlementaire, sans rien céder sur l'unité nationale, sans la laisser mettre en péril. au nom de cette unité nationale, affaiblir les garanties fondamentales. Trouvons un équilibre entre le maintien de l'ordre public et la sauvegarde de nos droits et libertés. La voie est étroite ; elle ne saurait en tout cas être celle d'une application rampante L'instauration d'un nouveau régime d'état d'urgence sanitaire sera pour nous une épreuve. L'état d'urgence sanitaire, tel qu'il est envisagé par le Gouvernement, diverge du régime d'état d'urgence issu de la loi du 3 avril 1955, que nous connaissons trop bien, hélas

n'aient de comptes à rendre à la représentation nationale. Les modalités d'entrée en vigueur de ce nouvel état d'urgence ne permettront pas au Parlement de le valider, ni même d'en débattre ou d'avoir simplement connaissance des mesures prises après son déclenchement. Le Gouvernement usera de ses pouvoirs exorbitants sans contrôle du Parlement, lequel sera simplement invité à dire « oui » ou « non » au déclenchement de l'état d'urgence sanitaire, sans rien savoir de son contenu

Pourtant, si l'on peut réunir quatre commissions cette semaine, il devrait être possible de mettre en place une commission spéciale de suivi capable de voter, au fil de l'eau, les mesures législatives nécessaires. C'est notre capacité de réaction qui est ici en cause : quelles que soient les mesures de confinement, nous montrons aujourd'hui que nous sommes capables de servir notre pays en conscience. Il nous appartient de résister à la tentation d'instituer des exceptions aux régimes d'exception. Dans ce cadre, monsieur le Premier ministre,

Une définition trop générale du champ d'application de la loi encourage à la prise d'innombrables mesures, favorise des pratiques variables et des marges d'appréciation illimitées. Il faudra encadrer celles-ci ; ce sera aussi notre travail.

le même niveau de contrôle de l'action gouvernementale que ce qui est prévu par la loi de 1955. Monsieur le Premier ministre, ce sont là les exigences minimales de la démocratie représentative dans le cadre d'un régime exceptionnel. Nous Nous assumons la situation exceptionnelle que vit notre pays, sans esprit de polémique, mais avec exigence et vigilance. Après le drame que nous vivons aujourd'hui, la France se redressera : c'est pour cela, mes chers collègues, que nous sommes fiers de la servir.

Monsieur le président, monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, les Français sont soumis depuis trois jours à des mesures lourdes, mais vitales. Confinés chez eux, ils ont suivi avec attention les prises de parole du Président de la République. Nos concitoyens respectent l'arsenal des mesures déployées par le Gouvernement pour protéger leur santé, assurer leur sécurité, maintenir leur emploi et garantir leur vote. L'urgence et la gravité de la situation nous réunissent aujourd'hui dans cet hémicycle pour transcrire dans la loi les annonces faites à nos concitoyens et à nos élus. En tant que parlementaires, nous devons permettre l'inscription dans notre législation et l'application dans les faits de ces mesures d'urgence. S'il est difficile d'imaginer dès aujourd'hui toutes les conséquences qu'aura la pandémie dans les jours, les semaines, et les mois qui viennent, nous devons tout de même nous y employer. Nous devons élaborer le cadre législatif d'un nouvel état d'urgence sanitaire pour les Français, tout en veillant à ne pas empiéter sur leurs droits. Les interdictions en vigueur concernant la liberté d'aller et de venir, la liberté de réunion ou la liberté d'entreprendre sont, dans ce texte, circonscrites dans le temps et dans l'espace. Pour garantir le contrôle parlementaire de l'action du Gouvernement, même dans des circonstances exceptionnelles où l'unité nationale doit prévaloir, l'Assemblée nationale et le Sénat doivent être informés sans délai des mesures prises pendant cet état d'urgence. Le Parlement est seul habilité à proroger, le cas échéant, l'état d'urgence sanitaire.

Nous devons tenter de remédier efficacement aux effets que la crise pourrait avoir sur notre économie et ses acteurs. Soutien à la trésorerie, aide à l'activité partielle, report du paiement des loyers et limitation des cessations d'activité et des licenciements sont essentiels si nous voulons garantir la survie de nos entreprises, en particulier de nos TPE et PME, qui constituent 99 % de notre tissu économique. J'ai défendu en commission, ce matin, un amendement visant à adapter le dispositif prévu en cas de catastrophe naturelle au régime d'urgence sanitaire, de manière à permettre aux départements de soutenir les entreprises. Je me réjouis que le Gouvernement ait été sensible à cette proposition et qu'il se soit engagé à la mettre en oeuvre par ordonnance. Nous devons aussi anticiper l'impact que la mise en suspens de notre vie quotidienne pourrait avoir sur les demandes de titres de séjour, les questions prioritaires de constitutionnalité, prioritaires de constitutionnalité, le nombre d'enfants pouvant être gardés par un même assistant maternel agréé ou le respect des horaires de travail. Les restrictions imposées en la matière par la loi ne pouvant être respectées, les mesures appropriées ont été intégrées à ce projet de loi. La nécessité d'agir vite et de manière proportionnée, dans chaque domaine de la vie économique et sociale de notre pays, doit faire loi, dans le respect du cadre de notre démocratie : c'est aussi une priorité. Ce projet de loi contient également des dispositions devenues indispensables à la réorganisation démocratique de nos assemblées locales. Nous devons asseoir les bases d'un pouvoir exécutif local stable, capable d'accompagner nos administrés en ces temps difficiles. Le combat contre le Covid-19 ne pourra se faire sans nos élus de proximité, comme je l'ai exprimé tout à l'heure à l'occasion de ma J'ai participé, au nom du président de mon groupe, à la prise de la décision que vient d'annoncer M. le Premier ministre, que je soutiens pleinement dans cette démarche. Oui, il nous faut reporter l'installation des conseils municipaux par conséquent, prolonger les mandats des élus de 2014 jusqu'à la fin du confinement. Nous reprendrons alors l'installation des nouveaux conseils municipaux.

Il nous faut également entériner les mesures visant à préserver le fonctionnement des syndicats de communes et des syndicats mixtes. En revanche, je suis farouchement opposée à ce que nous obligions les candidats au second tour

l'expérience dans laquelle nous sommes engagés et sur laquelle les pouvoirs publics continuent de réfléchir, adopter un régime original qui n'a pas à être calqué sur l'état d'urgence sécuritaire.

Je ne mentionnerai que brièvement le débat sur l'adaptation de nos collectivités territoriales à ce moment de crise. Nous constatons une

Nous devons aménager les procédures pour le cas où cette crise serait plus longue que prévu, de manière à assurer la continuité légale du fonctionnement de nos collectivités territoriales, soutiens essentiels de l'action de l'État en période de crise, comme on l'a vu dès les premiers jours. Je veux, en conclusion, Je veux, en conclusion, saluer le climat de compréhension et d'unité nationale qui a inspiré l'essentiel de notre débat. Nous devons nous placer à cette hauteur, en sachant que nous aurons,

non à la discorde ou à la critique politique. L'heure est à la reconnaissance envers tous ceux qui sont en première ligne, au contact des malades, et qui se battent souvent avec des moyens insuffisants,

le plan financier, les dépenses seront énormes, mais il faut les engager. C'est la valse des milliards ! Peut-être serait-il utile de prévoir la possibilité d'utiliser les comptes d'heures stockées, voire les RTT, pour être en mesure de relancer plus fortement la machine

monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes réunis cet après-midi dans les circonstances difficiles que vous connaissez. Alors que l'épidémie du nouveau coronavirus a connu une forte progression dans notre pays durant ces derniers jours, le chef de l'État et le Gouvernement ont proposé une série de mesures d'une ampleur considérable, visant à maîtriser la situation et à ralentir la progression du virus. Nous discutons aujourd'hui de leur concrétisation législative. Avant d'évoquer le contenu de ces mesures, je tiens à rendre hommage à ceux qui, face à la maladie, sont depuis le début au premier rang. Je parle bien évidemment de l'ensemble des personnels soignants, ainsi que des membres des forces de sécurité. S'il est vrai, comme l'a affirmé le Président de la République, que nous sommes en guerre, alors ce sont eux les soldats du front les plus exposés, dont le dévouement dans l'assistance aux malades et la mise en place des mesures de sécurité sanitaire doivent nous inspirer et nous inciter à agir avec solidarité et responsabilité. Avec solidarité, parce qu'en ces heures éprouvantes l'entraide et l'assistance à son prochain sont d'autant plus essentielles. Elles permettront de protéger les membres les plus fragiles de notre société, ceux qui, en raison de leur âge ou de leur

l'importance et l'efficacité et, par conséquent, de mettre en danger des vies humaines. Il faut que chacun prenne ses responsabilités, avec sérieux et sans pessimisme. Agissons donc avec discernement, que ce soit en respectant les préconisations des autorités sanitaires ou en évitant de colporter des informations douteuses. Venons-en au fond des textes présentés. Il s'agit d'un ensemble de mesures destinées à aménager la vie publique, économique et sociale des prochains mois, au regard des perturbations

certaines de ces mesures sont discutables. Il en est ainsi de la fixation de la date de dépôt des listes pour le second tour. Il serait préférable de la fixer explicitement au plus tôt, au lieu de la remettre au deuxième lundi précédant une date de scrutin encore incertaine, en faisant ainsi sortir davantage encore le déroulement de ces élections du droit commun. L'existence de conseils municipaux incomplètement élus présente également certains enjeux. Le texte du Gouvernement prévoit que, dans les petites communes, puisse être élu ce qui s'apparente à un « maire temporaire ». Cette solution est susceptible de soulever des interrogations sur la sincérité du second tour du scrutin. En l'état actuel du droit, le maire sortant continue d'assurer après le premier tour certaines fonctions de gestion des affaires courantes et des urgences. N'est-il pas plus simple de prolonger le mandat des conseillers municipaux sortants et de prévoir le maintien de cette situation jusqu'à ce qu'un nouveau conseil municipal La situation des communautés de communes est également complexe. Elles voient cohabiter des communes dotées d'un conseil municipal avec d'autres où celui-ci est incomplet. Là aussi, le Gouvernement semble privilégier la solution d'un « exécutif

afin de rendre possible un fonctionnement à distance. Faisons encore plus confiance à nos élus locaux en ces temps de crise. Enfin, le projet de loi ordinaire prévoit la création d'un état d'urgence sanitaire, reprenant de manière transparente certains des modes la loi de 1955 relative à l'état d'urgence. Il s'agit là, potentiellement, d'un outil puissant de lutte contre l'épidémie. Par certains aspects, ce régime est même plus exigeant que celui de l'état d'urgence « ordinaire

et du bilan viendra, l'heure est aujourd'hui à la cohésion nationale, à la responsabilité et à la solidarité. Il s'agit, pour le Parlement, de donner au Gouvernement les moyens de gérer cette crise et d'éviter une paralysie des collectivités territoriales. Je salue l'esprit de responsabilité des différents groupes politiques et du président-rapporteur de la commission des lois, qui, en dialogue avec le Gouvernement, proposent des dispositions de nature à répondre à l'urgence, tout en veillant scrupuleusement

avec dilatation du délai pour la tenue du second tour, mais maintien du dépôt des listes dans la foulée du premier tour, et à la modification des délais et des conditions de quorum et de procuration.

le groupe Union Centriste se tiendra à vos côtés et ne faillira pas à son devoir. En effet, notre pays, malgré la noirceur de certains comportements constatés ces dernières semaines, prouve, par l'engagement admirable de ceux que vous avez appelés, monsieur le Premier ministre, les « soldats du quotidien », sa capacité à tenir, à faire face, calme et droit, comme aime à le dire le premier d'entre nous ... Nous avons rendu hommage à la mobilisation des maires et de leurs services. D'ailleurs, nous proposerons un amendement sur le délai de carence des personnels municipaux. Je salue aussi les autres « essentiels », ceux qui soignent, mais aussi tous ceux qui nourrissent la France, car tous participent à la cohésion sociale, si fragile en ce temps de crise. temps de crise. L'urgence de procurer les équipements de protection nécessaires aux personnels de santé s'impose, bien entendu, mais il est tout aussi prioritaire de protéger ceux qui nous nourrissent,

monsieur le Premier ministre, messieurs les ministres, mes chers collègues, rien ne sera plus jamais comme avant. La situation que nous vivons est tout à fait inédite depuis plusieurs générations une crise sanitaire mondiale entraînant la prise de mesures privatives de liberté, nécessaires pour contenir l'épidémie, un système hospitalier submergé par la gravité de la maladie et, au premier plan de ce cataclysme, un arrêt brutal de notre économie et de l'économie mondiale. la fin d'un monde pour les enfants gâtés que nous étions ! Plus que jamais, l'heure est à la responsabilité collective et au consensus. C'est dans ces circonstances exceptionnelles que le Parlement se réunit pour examiner deux projets de loi.

Comment accompagner cette crise économique dans le temps ? À la période de confinement succédera la reprise d'une vie normale, mais les entreprises seront durablement affectées. Les conséquences de la crise sur la trésorerie, la consommation, l'investissement se feront ressentir dans la durée. Comment mettre en oeuvre les différentes les mesures économiques de façon simple, sans lourdeurs administratives, pour que les entreprises touchées par la crise en bénéficient rapidement ? Quelle Quelle coordination est mise en place avec les autres pays de l'Union européenne ? Le Conseil européen a d'ores et déjà annoncé un plan de 25 milliards d'euros, mais, on l'a vu en 2008, une coordination des différentes politiques nationales est nécessaire pour résister à une crise mondiale. Quel modèle économique voulons-nous pour demain ? Il faudra peut-être envisager la relocalisation de certaines activités, accompagner les entreprises dans ce sens, renforcer les différents modèles agricoles ... Nous devrons nécessairement engager une réflexion de fond. Cette crise sans précédent doit nous inciter à créer un nouveau modèle économique et agricole. Sur la forme, les mesures économiques sont inscrites dans des habilitations très larges données au Gouvernement pour légiférer par voie d'ordonnances. Si, au Sénat, nous ne sommes généralement pas très favorables aux ordonnances, car elles dessaisissent le Parlement de ses prérogatives, les circonstances exceptionnelles et l'urgence d'agir vite dans le domaine économique justifient entièrement que l'on y recoure. nous investirons bien entendu pleinement dans notre mission de contrôle de l'action du Gouvernement. Sophie Primas a notamment annoncé la mise en place d'une cellule de veille au sein de la commission des affaires économiques pour suivre la mise en oeuvre du plan du Gouvernement et faire remonter les difficultés et problématiques spécifiques de chaque secteur d'activité. Sur le fond, les mesures du plan d'urgence, qui ont pour finalité de limiter les cessations d'activité d'entreprises, quel qu'en soit le statut- cela est très important -, seront provisoires. Elles concerneront le soutien à la trésorerie et l'attribution d'aides directes ou indirectes aux entreprises dont la viabilité est mise en cause, notamment grâce à la mise en place d'un fonds de solidarité pour les TPE et les les TPE et les indépendants, dont le financement sera partagé avec les collectivités, la modification des obligations des entreprises à l'égard de leurs clients et de leurs fournisseurs, notamment en termes de délais, de pénalités et de nature des contreparties, le report ou l'étalement du paiement des loyers, des factures d'eau, d'électricité et de gaz afférents aux locaux pour les très petites entreprises, dont l'activité est affectée par les mesures prises pour limiter la propagation du virus, il sera demandé aux fournisseurs de renoncer aux pénalités financières et aux suspensions ou réductions de fourniture, en cas de non-paiement de ces factures l'adaptation des dispositions relatives à l'organisation de la Banque publique d'investissement, afin de renforcer sa capacité à accorder des garanties. Toutes ces mesures seront complétées par des dispositions relevant du code du travail. Je pense notamment à la prise en charge de nouvelles catégories de bénéficiaires au titre du chômage partiel. C'est parce que nous, sénateurs, sommes des relais essentiels de nos territoires que nous savons que tout cela va indéniablement dans le bon sens. Beaucoup de questions restent néanmoins en suspens, et j'espère que le Gouvernement pourra nous éclairer.

Quelle garantie a-t-on que le Gouvernement entendra cette revendication, monsieur le Premier ministre ? de leur chiffre d'affaires ces trois prochains mois ? Est-il envisagé que les banques ne facturent pas les frais de découvert et les agios ? Plus que jamais, les entreprises ont besoin de nous tous à leurs côtés ; elles ont besoin que nous agissions vite dans ces circonstances exceptionnelles. Elles peuvent compter sur l'engagement du groupe Les Républicains.

nous devons raffermir le cadre juridique dans lequel s'inscrivent les mesures que nous avons été conduits à prendre et que nous devrons prendre dans les jours et les semaines à venir.

viens aux remarques relatives aux dispositions concernant les élections municipales. Je salue le travail de la commission des lois, qui a su trouver des solutions à des questions que nous aurions pensé

dans des secteurs spécifiques. J'ai d'ailleurs précisé que, dans cet océan d'incertitudes, nous étions collectivement incapables de dresser la liste de toutes les mesures de nature législative qu'il nous sera nécessaire de prendre rapidement pour aider les entreprises, les salariés, les indépendants.